30 %, tandis que celui des crédits de paiement augmente de 50 %. Si l'on enlève l'opération particulière du programme 365, qui a trait à la recapitalisation de

Le nouveau programme 365, quant à lui, a pour objet la recapitalisation, à hauteur de 953 millions d'euros, de l'Agence française de développement, afin de respecter des règles prudentielles qui s'imposent à l'ensemble des établissements financiers et bancaires.

après l'intervention de mon collègue Michel Canevet sur les crédits prévus pour 2021, j'en viens à l'appréciation de la politique d'aide publique au développement mise en oeuvre par la France depuis plusieurs années. En 2021, les crédits de la mission poursuivent leur trajectoire haussière. En effet, l'aide publique au développement de la France a amorcé une augmentation depuis 2015, et elle a dépassé le montant de 10 milliards d'euros en 2017. En 2019, elle devrait atteindre 10,9 milliards d'euros. Cette augmentation a permis à la France de maintenir son rang, à défaut d'améliorer son classement, parmi les principaux contributeurs de l'OCDE, Ainsi, en 2019, la France reste le cinquième pourvoyeur d'aide publique au développement en volume, après les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Le pilotage de cette politique publique a fait l'objet de critiques nourries depuis plusieurs années. En effet, fortement interministérielle, la politique d'aide publique au développement apparaît éclatée, en raison des multiples instruments budgétaires qu'elle convoque et de l'intervention de plusieurs acteurs publics, tels que le ministère des affaires étrangères, le ministère de l'économie et l'Agence française de développement. Les auditions menées nous ont toutefois confortés dans l'idée que l'amélioration du pilotage était désormais une priorité des ministères en charge de ce budget. Dans cette perspective, les conclusions du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le Cicid, de février 2018 ont permis de fixer les priorités politiques et géographiques de notre aide publique au développement. Ce cadrage doit maintenant être confirmé au niveau législatif par une loi de programmation, qui devra redéfinir l'architecture du pilotage de la politique de développement. Annoncé à plusieurs reprises, le projet de loi n'a toujours pas été présenté en conseil des ministres Ces reports successifs deviennent préoccupants, dans la mesure où ce texte a vocation à constituer la boussole de l'aide publique au développement pour les prochaines années. Il nous reviendra de définir les dispositions législatives permettant d'encadrer le plus efficacement possible le fonctionnement de cette politique publique, qui constitue un instrument incontournable de l'action extérieure de l'État et du rayonnement

dans l'appétence de la France pour les prêts, au détriment des dons, nous encourageant ainsi à investir dans des pays à revenus intermédiaires, qui, comme tels, peuvent rembourser les emprunts. Plus généralement, ce constat nous conduit à nous interroger sur la stratégie mise en oeuvre à l'égard des « très grands émergents », pour lesquels l'accès à l'aide publique internationale n'apparaît plus comme une nécessité. En tout état de cause, les interventions dans ces pays doivent s'inscrire dans une parfaite adéquation

que multilatéral, avec l'initiative de suspension du service de la dette. Face à la crise sanitaire, les priorités de long terme ont néanmoins été préservées, telles que les soutiens au climat, à l'éducation ou à la lutte contre les « fragilités » et les « vulnérabilités » de certains pays. la dégradation des finances publiques renforce nos exigences en matière de transparence et d'évaluation de l'efficacité de cette politique publique. Ainsi, des dispositions permettant une évaluation indépendante devraient figurer dans le projet de loi à venir. loi à venir. J'en viens à l'examen de l'article 53 du projet de loi de finances rattaché à la mission. Il s'agit d'autoriser l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Aide publique au développement » vont connaître une nouvelle progression en 2021. En particulier, les crédits de paiement attribués à l'Agence française de développement, l'AFD, augmenteront de 154 millions d'euros, soit de 26 %. Sur cette toile de fond plutôt positive, j'évoquerai néanmoins deux préoccupations importantes de notre commission. Premièrement, comme l'a confirmé la Cour des comptes au début de l'année, l'AFD souffre d'un défaut de pilotage. L'Agence s'est trop autonomisée, devenant une sorte de « super-banque » tournée vers les grands émergents. Sa puissance de frappe, de l'ordre de 14 milliards d'euros, explique en partie cette évolution, face à une tutelle qui, elle, a dû au contraire se serrer la ceinture.

Il faut également simplifier l'empilement d'instances qui prétendent encadrer l'AFD et renforcer les capacités de la direction générale de la mondialisation, du développement et des Surtout, une double étape doit désormais être rapidement franchie pour consolider cette reprise en main, en commençant par la présentation du nouveau contrat d'objectifs et de moyens aux deux assemblées-

Cette loi aura pour ambition, nous l'espérons, une réforme de la politique d'aide au développement ; elle doit notamment prévoir la mise en place d'une commission d'évaluation véritablement indépendante- nous y veillerons.

fonds propres. Nous souhaitons, du reste, que toute éventuelle mesure de recapitalisation fasse l'objet de contreparties importantes de la part de l'Agence : maîtrise des charges, voire désengagement partiel des grands pays émergents, tels que la Chine ou la Turquie. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire où en est la réflexion sur un tel projet de recapitalisation ? D'autre part, la majorité des pays africains frôlent le surendettement. L'Agence ne pourra bientôt plus leur prêter. Au total, il sera donc nécessaire d'apporter de profonds changements au fonctionnement de l'AFD. Nous avons, vous l'avez compris, des réserves importantes sur ce budget publique au développement bénéficie aujourd'hui aux pays les moins avancés ; un renforcement du pilotage de l'AFD est en cours, mais nous attendons des résultats ; quant à la loi d'orientation, elle ne nous a toujours pas été présentée. Compte tenu de l'augmentation des moyens alloués et eu égard aux perspectives que la future loi pourrait dessiner, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a cependant émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission.

le budget de l'aide publique au développement est en augmentation, ce qui nous permet de reprendre progressivement notre rang en la matière ; il nous faut nous en féliciter. Je formulerai quelques remarques, j'évoquerai de nouveau la question de l'affectation de la taxe sur les transactions financières, ou TTF. Celle-ci a été créée explicitement dans l'objectif d'alimenter l'aide publique au développement, l'idée étant d'y faire contribuer les gagnants de la mondialisation. son produit, qui est de 1,6 milliard d'euros en 2020, est fléché vers l'APD. Parallèlement, nous assistons à l'effondrement du produit de la taxe sur les billets d'avion. Ne serait-il pas cohérent de compenser cet effondrement par une augmentation de la part de TTF ? J'ai déposé un amendement d'appel en ce sens, mais j'ai eu le regret de constater que M. le ministre délégué aux comptes publics n'a pas souhaité ou n'a pas pu en débattre. Quelle est donc, monsieur le ministre, votre position sur cette proposition ?

À l'occasion du G7 de Biarritz, en août 2019, le Président de la République a annoncé que la France doublerait sa contribution, ce qui est une bonne chose. Or, si le Fonds vert a levé au total 10,3 milliards de dollars de ressources, la part américaine de 2 milliards d'euros n'a toujours pas été versée.

À cette occasion, notre pays devrait travailler à ce que la part visant à l'adaptation au changement climatique soit rééquilibrée par rapport à la part visant à l'atténuation dudit changement. En effet, 25 % seulement des projets visent l'adaptation,

que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

La France est l'un des principaux acteurs en matière d'aide publique au développement. En 2019, elle conservait son cinquième rang mondial avec 12,2 milliards de dollars en volume, derrière les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Aujourd'hui, l'enjeu pour la France est de tenir son rang face aux autres puissances européennes et mondiales. Après cinq ans de baisse entre 2010 et 2015, l'aide publique au développement (APD) est la politique publique qui enregistre la plus forte hausse relative pour l'année 2021 plus 17 %. C'est un effort sans précédent en faveur de la solidarité internationale. Certes, cet effort pourrait être considéré comme peu prioritaire face à la somme de nos problèmes nationaux, mais n'oublions pas que toutes les économies sont aujourd'hui liées entre elles, dans un contexte où les dettes publiques s'alourdissent considérablement. Je tiens à saluer le travail de mes collègues Hugues Saury et Rachid Temal, rapporteurs pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des

2 millions d'euros sont réservés au Forum Génération Égalité, qui se tiendra à Paris en 2021- c'est un symbole fort pour les droits des femmes. Des fonds dédiés à l'aide humanitaire sont en hausse, avec 330 millions d'euros des efforts pour renforcer la part des dons sont maintenus. Enfin, dans ce contexte de pandémie, 60 millions d'euros sont consacrés au secteur de la santé dans le programme 110. Pourtant, l'an dernier, des doutes avaient été exprimés dans cet hémicycle sur le pilotage et la transparence de l'APD. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous avez fait de la recherche d'un meilleur pilotage politique une priorité. Nous notons avec satisfaction le renforcement du rôle de l'administration centrale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour mieux encadrer la diplomatie du développement, et la réactivation du conseil d'orientation stratégique de l'Agence française de développement, l'AFD. Le programme 365 vise à renforcer les fonds propres de l'AFD pour pérenniser les ressources et reboucler le circuit financier. De nouveau, l'APD ne doit pas être une politique isolée. La réforme des modèles économiques des acteurs du secteur pour intégrer les financements croisés de l'Union européenne et de la Banque mondiale va dans le bon sens. Depuis l'an dernier, le projet d'une taxe sur les transactions financières européennes poursuit son développement et, nous l'espérons vivement, permettra demain d'abonder l'APD. Depuis toujours, les restructurations et annulations de dette s'étalent sur plusieurs années, sans dommage majeur pour notre propre balance budgétaire. Surtout, elles sont nécessaires pour éviter que des pays ne soient en faillite, en pleine crise du covid, ce qui endommagerait leur capacité ultérieure à rembourser qui que ce soit. Tous les rapports ont été adoptés dans les différentes commissions sans modification. Bien sûr, le projet de relocalisation du siège social de l'AFD mérite notre attention et appelle notre vigilance. Toutefois, j'espère que ces garanties sauront apporter une réponse aux doutes exprimés l'an dernier sur ce budget. Au vu du caractère vital de l'aide publique au développement et de la responsabilité que nous avons en tant que nation, le groupe RDPI votera favorablement les crédits de cette mission.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, une fois encore, nous allons adopter les crédits de la mission « Aide publique au développement » sans le cadrage maintes fois promis- ce sera peut-être encore le cas ce soir -, mais toujours pas mis en oeuvre, d'une loi de programmation pluriannuelle de l'aide publique au développement. C'est d'autant plus problématique qu'aux enjeux structurels sur l'absence d'un ministre dédié, sur les montants de cette aide publique, sur sa conception, sur ses critères sur la transparence de sa mise en oeuvre s'ajoutent désormais les effets durables, structurants et aggravants en termes d'inégalités de la pandémie sur des pays destinataires déjà bien fragiles. C'était donc, à l'heure de toutes les urgences, le moment de présenter cette loi de programmation. Or nous n'y sommes toujours pas. Cela en dit long sur les retards pris et sur la sous-estimation des enjeux ! Quoi qu'en disent les chiffres annoncés, nous sommes très loin d'être au niveau, en termes tant de montants que de réorientation stratégique de cette aide publique. Pour cette année encore, les prêts représentent l'écrasante majorité de l'activité de l'AFD : comparés aux 16 % en moyenne des autres pays du Comité d'aide au développement, c'est peu de dire que nous devons poursuivre et accélérer une profonde réorientation. La domination des prêts a des conséquences fortes. Elle oriente une part importante de nos aides vers les pays les plus solvables, au détriment des plus fragiles qui devraient avoir la priorité, alors même que, pour la première fois en vingt ans, l'extrême pauvreté reprend sa progression dans le monde.

au même titre que l'amplification d'un continuum entre développement et sécurité, l'intégration dans l'APD des questions migratoires ou la récurrence de l'aide conditionnée, dont les critères sont tous centrés sur une prétendue et discutable « défense de nos intérêts » et non sur les véritables enjeux du développement tels qu'ils sont définis par l'ONU. Le pré-projet de loi de programmation, rédigé bien avant que n'explosent les besoins liés la crise sanitaire, tablait sur une mission « Aide publique au développement » pour 2021 entre 3,9 milliards et 4 milliards d'euros, auxquels il fallait ajouter 838 millions d'euros alors prévus d'affectation de taxes. Nous sommes, il est vrai, aujourd'hui au-dessus

TSBA. La France, cinquième puissance économique du monde, prévoit de participer à hauteur de 1 % à l'aide d'urgence demandée par les Nations unies pour les pays les plus pauvres, qui subissent de plein fouet toutes les crises. La coordination des ONG estime, quant à elle, que la France pourrait d'ores et déjà mobiliser des sommes beaucoup plus importantes, soit près de 15 milliards d'euros de plus, notamment grâce à une autre politique de gestion de la dette et surtout à une augmentation plus audacieuse des taxes et ressources dédiées à l'APD.

de nombreux autres pays, la France est elle-même sinistrée. Avec la pandémie, son économie- notre économie -a été durement touchée : le chômage repart à la hausse, des entreprises ont mis la clé sous la porte et la pauvreté augmente sur notre territoire. Cependant, nous examinons aujourd'hui les crédits destinés à aider d'autres pays à se développer, en leur faisant moins de prêts et plus de dons. Alors que la situation économique de notre pays est historiquement mauvaise, certains pourraient avoir du mal à comprendre que la France cherche cette année encore à atteindre ses objectifs en matière d'aide au développement. La formule des années 1960 « La Corrèze avant le Zambèze » pourrait ainsi revenir au goût du jour et Territoires considère cependant que la poursuite de l'action de la France en la matière est primordiale. À deux principaux égards, l'aide publique au développement est un outil précieux dans les relations internationales. D'une part, l'interdépendance des économies nationales n'est plus à démontrer. Un pays qui se développe grâce à la France est un partenaire économique. En renforçant ses infrastructures et en améliorant le niveau de vie de sa population, ce pays développe des conditions d'échanges propices au renforcement des liens institutionnels et aux opportunités entrepreneuriales avec la France. Dans une économie mondialisée, aider au développement des autres, c'est indirectement favoriser son

Les zones les plus instables sont souvent celles où le développement est le plus faible, en particulier lorsque l'État n'a pas les moyens de mettre en place une instruction publique. En Afrique, plus particulièrement au Burkina Faso, près de 2 300 établissements ont fermé fermé à cause du terrorisme. C'est dans un tel contexte que l'aide au développement est primordiale afin de lutter contre le risque d'embrigadement des enfants dans des écoles du terrorisme. Pour éviter la création de zones de non-droit dans des États qui connaissent une certaine instabilité, il est essentiel de les accompagner dans un développement homogène de leur territoire. Le développement contribue ainsi à la résolution politique de conflits qui nous concernent. C'est notamment le cas des pays de la bande sahélo-saharienne. Pour avoir le meilleur effet, l'aide doit être concentrée sur les pays qui en ont le plus besoin. À cet égard, nous comprenons et nous soutenons le changement de logique consistant à privilégier les subventions et les dons plutôt que les prêts. L'aide est souvent plus cruellement nécessaire aux pays qui n'ont pas la capacité de rembourser. La France avait jusqu'à présent préféré accorder une aide sous forme de prêts pour des raisons évidentes d'allégement des coûts. Cela a néanmoins conduit à diriger des aides vers des pays qui ne semblent pas être les plus prioritaires. Si le remboursement des prêts que la France accorde à la Chine paie le salaire du directeur de l'Agence française de développement, il n'en est pas moins difficile de justifier que Pékin, capitale de la deuxième puissance mondiale, puisse avoir besoin de l'aide Nous devons nous assurer que l'argent consacré à l'aide publique parvient effectivement aux projets choisis par la France. Dirigée vers les pays qui en ont le plus besoin, majoritairement sous forme de subventions, l'aide publique au développement devra en outre faire l'objet de contrôles d'autant plus étroits.

Dans un climat national où la pauvreté sera de plus en plus apparente, nous devons être très vigilants sur toute dépense ostentatoire. Veuillez conclure, mon cher collègue. Il convient que ces charges de fonctionnement soient les plus faibles possible afin que chaque euro dépensé contribue avant tout à lutter contre la pauvreté et les inégalités dans le monde.

Madame la présidente, monsieur le ministre, confirmant la trajectoire engagée en 2018 et les promesses présidentielles, la mission « Aide publique au développement » est en hausse de près de 50 % pour atteindre 4,9 milliards d'euros en crédits de paiement. Cette augmentation s'explique toutefois en très grande partie par un nouveau programme de recapitalisation de l'Agence française de développement, qui vise principalement à se conformer qui vise principalement à se conformer aux nouvelles règles prudentielles européennes. Il n'en reste pas moins que c'est une hausse que je tiens à saluer, d'autant qu'elle permet de se rapprocher de l'objectif de 0,55 % du RNB dédié à l'aide publique au développement à l'horizon de 2022. Toutefois, ne nous méprenons pas, cette hausse n'est en réalité qu'un rattrapage. En 2010, 0,5 % du RNB était consacré à l'aide publique au développement. Aussi, la France est toujours loin de l'objectif de 0,7 % auquel elle s'est engagée dans une résolution de l'ONU, en 1970. L'augmentation des budgets n'est pas encore suffisante pour que l'aide au développement de la France joue le rôle qui doit être le sien. Un récent rapport d'Oxfam intitulé « 50 ans de promesses non tenues » chiffre à 5 000 milliards d'euros sur cinquante ans les sommes non versées. La pandémie accentue par ailleurs les besoins en termes de financement. Alors que plus de 100 millions de personnes risquent de tomber dans l'extrême pauvreté, l'ONU évalue à 500 milliards d'euros les besoins supplémentaires pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique. Pour la France, au regard de son poids dans l'économie mondiale, cela représenterait 14,5 milliards d'euros supplémentaires. Nous n'y sommes pas encore ... Au-delà de la recapitalisation de l'AFD- j'exprime au passage ma circonspection sur l'opération immobilière à plus de 800 millions d'euros prévue par

examine les chiffres dans le détail, la répartition des crédits de la mission soulève plusieurs interrogations. Je tiens tout d'abord, chers collègues, à appeler votre attention sur le grand paradoxe de l'aide publique au développement française : ce ne sont pas les dix-neuf pays considérés comme prioritaires qui bénéficient le plus de l'aide. Cette aberration

Plutôt que de contribuer financièrement à l'agrandissement des lignes de métro d'Istanbul, nous ferions mieux d'aider les pays prioritaires. D'après Jorge Moreira da Silva, chargé de la direction de la coopération pour le développement à l'OCDE, « le financement du développement durable des pays en développement risque de s'effondrer Il faut donc passer outre les règles prudentielles et aider les pays qui n'ont pas les moyens d'assurer leur transition énergétique. Sur les dix-neuf pays, dix-huit sont africains. Allouer les crédits destinés à la Chine à ces dix-huit pays permettrait d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Telle devrait être la vocation première de cette mission budgétaire. Enfin, il est essentiel de revenir sur la question des conditionnalités. Il serait inutile de conditionner l'aide publique au développement à des engagements en matière migratoire. Le but de l'aide publique au développement est que les pays bénéficiaires puissent s'ouvrir au monde de façon autonome. L'aide publique au développement ne doit pas devenir le pendant de la politique migratoire française. La prise en compte du taux de reconduite à la frontière n'aidera pas les pays bénéficiaires à relever les défis contemporains. Conditionner les aides à des clauses migratoires ne ferait que régler les manifestations du problème, En bref, nous examinons un budget habituel alors que nous sommes face à une crise exceptionnellement grave. Nous ne pouvons pas voter favorablement des crédits que même l'OCDE juge insuffisants.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un monde brutalement mis à l'arrêt par la pandémie de la covid-19, les aides tant privées que publiques en direction des pays pauvres sont fortement affectées : 700 milliards de dollars en moins selon une estimation de l'OCDE. Dans ce contexte difficile, malgré la crise économique et la dégradation des finances publiques que connaît notre pays, je salue l'action du Gouvernement, qui entend viser l'objectif de hausse continue du budget de l'aide publique au développement établi à 0,55 % de notre revenu national brut d'ici à 2022. Cet effort illustre l'attachement de la France à une politique qui est l'expression de ses valeurs de solidarité et d'humanisme. Je rappelle que notre pays est le cinquième pays pourvoyeur mondial d'aide publique au développement. Je rappelle également que la France a fortement appuyé l'initiative de suspension du service de la dette, l'ISSD, actée entre le Club de Paris et le G20 avant l'été. Cette politique est en outre un levier important de notre rayonnement international, en particulier quand elle s'exerce à travers une coopération bilatérale, qui donne une visibilité plus directe de nos actions sur le terrain. Aussi, je me réjouis de constater la confirmation de cette orientation dans ce projet de loi de finances. Je pense notamment à l'augmentation des moyens de l'Agence française de développement au titre des dons-projets et des dons-ONG. Je souligne enfin que la politique de développement est un instrument de diplomatie de la paix. Il est bien évident que la pauvreté nourrit l'instabilité et fait le lit des organisations criminelles ou terroristes. Mardi dernier, l'Union européenne s'est engagée à prêter 1,2 milliard d'euros à l'Afghanistan, tout en appelant les talibans à s'impliquer concrètement dans le processus de paix. À cet égard, il me semble que la conditionnalité des aides ne doit pas être un sujet tabou. Au-delà de ces trois axes, qui doivent continuer de mobiliser notre politique d'aide au développement, je souhaite évoquer quelques-unes des priorités qui me paraissent essentielles et dont, je l'espère, nous pourrons bientôt débattre dans le cadre du projet de loi de programmation tant attendu. En effet, les questionnements relatifs à l'orientation de l'aide publique au développement sont nombreux. Sur sa nature, je crois qu'un large consensus existe pour privilégier une politique de dons et de subventions plutôt que de prêts,

Sur l'orientation géographique, est-il bien opportun, dans les conditions politiques que nous connaissons, de reconduire notre soutien, notamment bilatéral, vers la Turquie ? Il a tout de même représenté 127 millions d'euros en 2018 Est-il bien raisonnable de continuer à aider la Chine, qui a enregistré une croissance de 4,9 % au troisième trimestre de 2020 ? En revanche, le Comité interministériel de coopération internationale et de développement de 2018

Ce débat est urgent, monsieur le ministre. Mes chers collègues, en attendant de redéfinir ensemble les contours de la politique de notre aide publique au développement et de répondre à toutes ces questions, le groupe RDSE votera les crédits de cette mission, qui envoient néanmoins des signaux positifs. La parole

après une baisse continue entre 2010 et 2015. Cette aide enregistre la plus forte hausse relative au budget de l'année 2021. Nous constatons sans équivoque qu'il s'agit d'un effort sans précédent en faveur de la solidarité internationale, effort qui s'inscrit dans le contexte économique actuel, qui pèse lourd sur nos finances publiques. Le groupe Union Centriste salue l'effort qui contribue à concrétiser l'engagement du Président de la République, celui de rattraper notre retard et d'atteindre 0,55 % du revenu national brut d'ici à 2022. Nous voterons donc les crédits de cette mission. Nous encourageons le fait que l'aide publique au développement et la réforme de la politique française de développement soient consacrées comme l'une des priorités du quinquennat. Il va sans dire que la réalisation de cet objectif est essentielle dans le contexte international, contexte où les crises successives et la montée des inégalités ne cessent de s'amplifier et où le multilatéralisme menace de se fissurer. De même, nous approuvons, bien entendu, que les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » respectent les conclusions du Conseil interministériel de la coopération et du développement de 2018. D'une part, la priorité géographique est respectée, avec 73 % des prêts qui doivent bénéficier à la région Afrique-Moyen-Orient. D'autre part, la priorité sectorielle est aussi constatée dans le contexte de crise sanitaire. Nous remarquons un soutien significatif en faveur de la santé mondiale, avec notamment 60 millions d'euros d'aides budgétaires globales dans le programme 110, 2 millions d'euros pour l'Institut Pasteur et plus de 10 millions d'euros en faveur du Fonds français Muskoka. Cependant, certains points appellent notre vigilance. Certaines évolutions relatives aux programmes 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » et 110 « Aide économique et financière au développement » sont à regretter. En effet, ces programmes resserrent les autorisations d'engagement puisqu'elles sont en baisse de 2,1 milliards d'euros, alors que les crédits de paiement sont en hausse de 1,6 milliard La pandémie a démontré la nécessité d'aller au-delà du renforcement du multilatéralisme. Pourtant, ce mouvement conduit à une baisse considérable de l'action Aide économique et financière multilatérale du programme 110. Cette diminution ne nous semble pas cohérente dans le contexte sanitaire que nous subissons. La raison et le sens commun voudraient que la France se maintienne et conserve sa capacité d'orientation des fonds gérés par les banques multilatérales de développement. Nous tenons à attirer votre attention sur un autre point. L'impact de la crise sanitaire dans l'aide publique au développement ne doit pas placer la situation d'urgence climatique au second rang de nos préoccupations. À titre d'exemple, le sud de l'île de Madagascar, que j'ai visité l'an dernier dans le cadre d'une mission interparlementaire, connaît aujourd'hui un épisode de sécheresse exceptionnel menaçant de famine plus d'un million de Malgaches. Cette Cette tragédie imminente nous rappelle l'importance d'annuler la dette des pays les plus vulnérables. Dans cet élan, des efforts ont été entrepris en concordance avec les engagements du Président de la République. Je fais référence à l'instauration d'un moratoire au service de la dette des pays les plus pauvres. Quant au Fonds monétaire international, il estime que des actions plus audacieuses sont nécessaires, comme la réduction des intérêts de la dette. En conclusion, l'action du Gouvernement gagnerait à être mieux hiérarchisée. Elle est cependant toujours définie par cet engagement originel, fixé en 1970 par l'Organisation des Nations unies : celui d'allouer au moins 0,70 % de notre richesse nationale brute à l'aide publique au développement. Vos efforts doivent tendre vers cet objectif. Nous plaçons donc nos espérances dans le projet de loi de programmation relatif à la politique de développement et à la lutte contre les inégalités mondiales, Aujourd'hui, l'actualité mondiale nous démontre plus que jamais à quel point l'aide publique au développement est cruciale. Plusieurs pays, plusieurs régions du monde sont en proie à des déséquilibres, qui laissent craindre, dans un futur proche, l'émergence de situations contraires à nos intérêts. Il est important de garder en mémoire que l'aide publique au développement, levier puissant de notre diplomatie, ne pourra répondre à ces défis communs que par la pérennisation d'une large solidarité internationale.

mais qui soulève toutefois deux inquiétudes et deux attentes. Notre première inquiétude concerne l'Agence française de développement. Les crédits de paiement délégués à l'AFD augmentent de 154 millions d'euros, soit 26 %. C'est beaucoup. Or, depuis plusieurs années, la forte augmentation des engagements de l'AFD a conduit la commission des affaires étrangères du Sénat à relever que le pilotage de cette agence était insuffisant. Cette analyse a été confirmée il y a quelques mois par un rapport de la Cour des comptes. Il est donc impératif que le nouveau contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD soit présenté aux assemblées et que la nouvelle convention-cadre entre l'État et l'AFD soit signée pour fixer le schéma stratégique, mais aussi démocratique, de notre aide publique au développement. il faut rééquilibrer la relation entre l'AFD et ses deux ministères de tutelle- le vôtre, monsieur le ministre, et le ministère des finances -, avec des objectifs clairs et bien définis. Il importe de pouvoir contrôler que les attentes des parlementaires et du Gouvernement Enfin, malgré certains progrès, la question d'une meilleure évaluation des résultats n'est pas résolue et la mise en place d'une commission indépendante d'évaluation paraît plus que jamais nécessaire.

Il est donc impératif de trouver des modalités de financement des pays les plus pauvres qui n'acculent pas, périodiquement, ces derniers à des situations d'endettement insoutenables. seconde inquiétude porte sur la disparition prochaine du Fonds européen de développement (FED), qui sera fusionné au sein d'un instrument unique de voisinage, de développement et de coopération avec pour conséquences probables une moindre focalisation sur l'Afrique subsaharienne et, à la demande de plusieurs pays d'Europe du Nord, une attribution plus importante de financement au pays des Balkans. Les nouveaux instruments comporteront sans doute une part de prêts réservés aux pays africains à revenus intermédiaires davantage qu'aux pays les plus pauvres du continent africain. Il faudra donc que la France veille à préserver la concordance de ces financements européens, auxquels elle va- comme toujours

concerne la taxe sur les transactions financières (TTF), dont plusieurs collègues ont déjà parlé. Cette année, son rendement sera plus élevé que prévu- tant mieux ! -, mais la part de cette taxe qui sera consacrée à l'aide publique au développement restera plafonnée, hélas, à 528 millions d'euros. Parallèlement, la taxe de solidarité sur les billets d'avion, qui alimente aussi le FSD, a vu son rendement s'effondrer du fait de la crise du transport aérien. Si cette diminution a été compensée par le budget général pour 2021, il serait souhaitable que le dynamisme de la TTF soit mis à profit pour assurer une compensation de la baisse de la TSBA. Enfin, en ce qui concerne la TTF, nous renouvelons, comme chaque année, notre souhait de voir augmenter son taux de 0,3 % à 0,5 % et allouer 50 % de ses recettes au FSD.

texte devrait permettre à la France de traduire de manière législative les engagements pris par notre pays pour respecter l'agenda 2030 de l'ONU et l'Accord de Paris sur le climat. L'avant-projet a été diffusé à la fin du

de loi en conseil des ministres, puis au Parlement. La société civile impliquée dans les problématiques du développement dans son ensemble dénonce le retard pris par la France et demande qu'une augmentation des crédits budgétaires soit inscrite dans la future loi. Elle

nos concitoyens. Il est véritablement temps de distinguer clairement ce qui relève de l'aide aux pays les plus pauvres et ce qui concerne plutôt le financement du développement durable dans les pays émergents. Ces deux objectifs sont tout à fait recommandables et nécessaires, mais ils ne se confondent pas. Très bien

les succès militaires que nos soldats y remportent chaque jour et que l'on peut saluer ne pourront aboutir à une paix durable que s'ils sont accompagnés par les succès du développement. Nous avons, sur ce plan, une véritable responsabilité.

l'encadrement d'une aide multilatérale encore trop peu transparente, l'intégration d'Expertise France dans le groupe AFD et la création d'une commission d'évaluation réellement indépendante.

des moyens consacrés à cette politique. Monsieur le ministre, cette nouvelle augmentation des crédits de l'APD, notamment des dons-projets, nous permettra de maintenir notre soutien à une Afrique d'ores et déjà ébranlée par les effets économiques du covid. Cette hausse a convaincu notre commission de soutenir

Le nouvel état d'un monde « covidé » cristallise plus que jamais les inégalités entre les pays et affecte durablement l'avenir des populations partout dans le monde, bouleversant encore davantage les équilibres géopolitiques. de mettre en place les dispositifs de production et d'acheminement d'aides d'urgence en matériels et équipements médicaux. Parallèlement, l'aide publique au développement est autant un vecteur de sécurité globale, reposant sur la sécurité alimentaire et énergétique, qu'un outil d'influence internationale et diplomatique. Cette influence intègre désormais la capacité d'un État à soigner, à gérer une pandémie sur son sol, au travers d'un système de santé et avec des ressources humaines, d'équipement et de recherche. À l'aune de ce contexte aux inédits multiples, vous comprendrez, monsieur le ministre, notre triple exigence. La première exigence concerne les objectifs de la politique française d'aide au développement. Quelles seront les priorités géographiques et stratégiques de l'APD en 2021 ? Quels pays bénéficieront des projets ?

Force est de constater que ces nouveaux impératifs rendent caduques les priorités de l'APD française définies dans le premier chapitre de la loi d'orientation et de programmation relative Une nouvelle loi, annoncée à grand renfort de communication en 2017, est toujours attendue. Il y a plus d'un an, les membres de la commission des affaires étrangères se sont mobilisés et ont commencé à travailler dans un esprit de proposition et de responsabilité. Monsieur le ministre, lors de votre audition au Sénat, le 3 novembre dernier, vous aviez déclaré qu'un projet de loi serait présenté à la fin du mois de novembre en conseil des ministres. Nous connaissons votre engagement personnel sur ce sujet et nous vous en remercions, mais nous désespérons d'une transmission de ce texte au Parlement avant la fin de l'année.

2021. Qu'en est-il en termes de volumes de crédits ? N'est-ce pas un effet mécanique résultant de la réduction du PIB liée à la crise et à l'annulation de la dette soudanaise ?

à l'équation de l'évaluation ? Logiquement alors, notre troisième exigence concerne la nature de l'aide, qui est indissociable de l'instauration d'un programme d'évaluation fondé sur la transparence. Nous ne pouvons que constater le fossé grandissant entre l'augmentation des montants dédiés à l'AFD et les carences de pilotage de ces fonds. Certes, l'Agence est une banque sous la tutelle de Bercy. pour autant une raison pour s'affranchir des recommandations des commissions des affaires étrangères et des finances du Sénat, ainsi que de la Cour des comptes, sur un problème aussi grave que le déficit de gouvernance, alors même que tous les acteurs du secteur privé déploient actuellement des efforts considérables pour répondre aux impératifs internationaux en termes de normes de gestion

500 mètres carrés dédiés aux espaces de réunion, au moment où les réunions internationales sont dématérialisées et où les grandes sociétés réduisent leurs parcs de bureaux parisiens ? À cet instant, je tiens à remercier les rapporteurs pour avis, Hugues Saury et Rachid Temal, qui ont alerté sur les déséquilibres inquiétants du modèle de prêt de l'AFD, lequel nécessite la mobilisation de fonds propres dont elle ne dispose pas. Monsieur le ministre, avant de conclure, j'aborderai un point important, la fiduciarisation de l'APD internationale. Les prises de participations dans des banques de développement, comme celles qui sont prises au sein de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, ou le sommet des banques publiques de développement, réuni à Paris le 12 novembre dernier, ne sauraient devenir les tendances lourdes de la politique de développement. L'ambition, l'expérience, la vision singulière de notre diplomatie, doivent redevenir la boussole d'une APD à la française. La parole est à M.

face aux défis globaux auxquels nous sommes confrontés, nous avons besoin d'une solidarité internationale accrue. C'est une question d'efficacité et de justice. C'est pourquoi, en accord avec le Président de la République et le Premier ministre, j'aurai l'honneur de présenter en conseil des ministres, le 16 décembre, ... Prochain effet ! ... puis devant la représentation nationale, le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

les sénateurs, une augmentation très significative- près de 17 % -, pour atteindre près de 2,5 milliards d'euros. nous permettra de poursuivre une trajectoire ascendante de l'APD, dans la perspective d'y consacrer 0,5 % de notre richesse nationale d'ici à 2022, conformément à l'engagement pris par le Président de la République. Sur ce point, je connais toutes les discussions

programme budgétaire dédié, qui a été créé pour doter l'AFD en capital à hauteur de 953 millions d'euros, afin de lui permettre de poursuivre son activité de prêt dans le respect de la réglementation bancaire. L'AFD est en effet soumise à deux ratios : un ratio « grands risques

et le ministre chargé de ce dossier, c'est-à-dire votre serviteur, examinent un second canal, passant par une dotation supplémentaire en capital de 500 millions d'euros qui serait proposée le moment venu par le Gouvernement. En tout état de cause, une telle dotation représenterait un nouvel effort financier important de la part de l'État pour soutenir l'AFD, dans un contexte budgétaire contraint, et devrait donc être assortie de contreparties très strictes pour l'Agence,

Par ailleurs, conformément aux orientations définies par le Président de la République, la composante bilatérale de l'aide publique au développement augmentera fortement en 2021, et ce d'abord au travers de la poursuite de la hausse des moyens alloués à l'AFD au titre de l'aide projet,

plus important poste budgétaire du programme, devant les crédits dédiés au FED. Dans cet ensemble, les fonds destinés à soutenir l'action de la société civile augmentent également : en 2021, les subventions dons-ONG

de l'aide bilatérale, le processus de programmation géographique et sectorielle des engagements de l'AFD est très clair : en 2019, ce sont 68 % des dons qui ont bénéficié aux dix-neuf pays prioritaires.

posé comme condition à mon soutien le respect de plusieurs exigences : d'une part, la neutralité du coût pour l'État- c'est le cas -, d'autre part, le droit de regard sur l'utilisation qui sera faite des 10 000 mètres carrés de surface excédentaire par rapport aux besoins du groupe AFD. Ce siège peut devenir

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Aide publique au développement », figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits. J'appelle en discussion

n° II-488 est retiré. Nous allons procéder au vote des crédits du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », figurant à l'état D. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite.

Merci